Leur impression est d’autant plus légitime que, lors de la mise en place du dispositif de collecte des DMTO, les grandes communes de plus de 5 000 habitants ont bénéficié immédiatement des ressources, tandis que les autres ont dû attendre une année supplémentaire en raison de la péréquation.

perçu sur le territoire des communes de moins de 5 000 habitants est versé à un fonds départemental de péréquation. Les ressources provenant de ce fonds sont ensuite réparties, l’année suivante, par le conseil départemental, entre les communes de moins de 5 000 habitants, selon trois critères légaux : l’importance de la population, le montant des dépenses d’équipement brut et l’effort fiscal de la collectivité bénéficiaire. concerne la répartition du fonds départemental, le conseil départemental devra en effet exclure une commune passée au dessus du seuil de 5 000 habitants en année de la répartition au titre de la même année ; c’est le cas de la commune de Saint Vit, que vous évoquez,

dès qu’une commune passe sous le seuil des 5 000 habitants en année , elle ne bénéficie plus de la taxe additionnelle au titre de cette année. En revanche, le conseil départemental est légitime à l’intégrer dans la répartition des ressources du fonds, à laquelle il procédera au titre de cette année, alors même que cette commune n’aura pas alimenté ce fonds l’année précédente.

avait été publiée avec un intitulé quasiment identique. Cette question s’adressait également au ministre de l’économie et des finances, lequel a publié une réponse le 14 avril 2022. Toutefois, la lecture de cette réponse laisse planer un doute quant à la correcte interprétation du terme « chronologique ». En effet, le ministre indique qu’une « commune ne peut pas lever la taxe locale sur la publicité extérieure en même temps que l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la redevance sur un même support, et réciproquement ». Il précise ensuite que « les textes ne prévoient pas de traitement spécifique en cas de double institution », ajoutant que, dès lors, « le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique

quelle est la juste interprétation du terme « chronologique » figurant dans la réponse du ministère ? Si « le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique », faut il prendre

le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un principe d’incompatibilité entre la perception d’une redevance d’occupation du domaine public et la taxe locale sur la publicité extérieure levée sur le même support. En effet, aux termes de l’article L. 2333 6 dudit code, « dès lors que la commune [ou son groupement] lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation du domaine public public ». Le législateur a ainsi entendu préserver l’occupant du domaine public de tout mécanisme qui conduirait à un double prélèvement, par la voie fiscale et domaniale, pour un même fait générateur : dès lors que la taxe est levée,

La France a devant elle un certain nombre d’échéances en matière de communications fixes et mobiles. En premier lieu, le dispositif dit du New Deal mobile, destiné depuis 2018 à garantir la couverture en téléphonie mobile de nos territoires, prendra fin en 2025. à son échéance, il manquera plusieurs milliers de pylônes pour assurer la couverture promise en 2018. En second lieu, le démantèlement du réseau de cuivre, entamé le 31 janvier dernier, devrait s’achever en 2030. Il mettra fin au réseau ADSL,

Cela aura également d’importantes conséquences, notamment pour les objets connectés : alarmes, dispositifs médicaux… J’ai donc trois questions simples. Tout d’abord, comment le Gouvernement prépare t il ces échéances ?

L’accord du New Deal mobile a été conclu en 2018 entre les opérateurs et l’État. Il a orienté l’effort des opérateurs vers la couverture du territoire, au moyen d’obligations de couverture inédites. Six ans après

Cette politique publique a coûté 3 milliards d’euros et s’est largement faite au profit des territoires ruraux, qui ont bénéficié du déploiement de 67 % des sites mobiles depuis le démarrage du New Deal.

Pour compléter cette couverture, les engagements pris au titre du New Deal participeront à la poursuite des déploiements au delà de l’année 2025, notamment pour la couverture en services mobiles à l’intérieur des véhicules sur la totalité des axes routiers prioritaires et la couverture des axes ferrés à l’intérieur des trains d’ici à 2030. Enfin, indépendamment du New Deal, des obligations de couverture contribueront également

ont changé le paysage fiscal pour les collectivités territoriales. Ce mouvement aurait dû s’accompagner d’une plus grande transparence de l’information fiscale et financière sur les ressources transférées. Or nous ne pouvons que déplorer le manque d’informations transmises. Les collectivités sont ainsi dans l’impossibilité de contrôler avec exactitude les montants attribués par l’État.

L’absence de transparence se remarque également dans le suivi de l’évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui concerne désormais directement les finances des collectivités, depuis la mise en place des mécanismes de compensation sur fraction de TVA.

et les collectivités, et cette confiance passe par une plus grande transparence. Les collectivités territoriales devraient pouvoir accéder à une information complète leur permettant de contrôler les modalités de calcul et vérifier ainsi la correcte et juste attribution des compensations dues par l’État.

? La parole est à Mme la secrétaire d’État. Monsieur le sénateur Grosvalet, en contrepartie de la suppression de la CVAE comme ressource locale, les collectivités bénéficient depuis 2023 d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette ressource donne lieu à actualisations annuelles, en fonction des prévisions des recettes de TVA. La DGFiP partage votre volonté d’accompagner au mieux les collectivités locales dans l’évaluation de leurs ressources fiscales ; pour cela, elle a mis en place plusieurs outils.

obligatoire est versé quotidiennement aux départements en fonction des cessions enregistrées, et les départements sont informés des versements par leurs comptables assignataires.

population vieillit. D’ici six ans, il y aura 49 % de Français âgés de 75 à 84 ans. Or la France n’est pas prête à répondre aux défis du vieillissement démographique. Aujourd’hui, le constat est partagé : la situation est catastrophique, pour reprendre les mots des professionnels du secteur du grand âge, qui ne cessent de lancer des alertes sur la situation, comme lors de la journée nationale du 24 septembre dernier.

Le précédent gouvernement n’a pas su consolider la situation financière de ces établissements : près de 80 % d’entre eux sont en situation de déficit. Ces structures ne disposent plus des moyens de mener à bien leur mission, pourtant essentielle dans la prise en charge des résidents,

date de 1873 – c’est la plus ancienne maison de retraite du département –, connaissent de grandes difficultés financières, malgré l’engagement et le sens du devoir du personnel. Ces difficultés entraînent des conséquences sur l’attractivité des établissements auprès des familles, mais aussi des emplois, du personnel soignant et d’accompagnement. Ma question porte donc sur la question du financement des structures d’accueil du secteur médico social. premier lieu, un an après la mise en place dans chaque département d’une commission dédiée au suivi et à l’examen de la situation financière des structures médico sociales en difficulté, quel est le bilan de ces commissions ?

Monsieur le sénateur Anglars, les crédits destinés aux établissements et services pour les personnes âgées ont augmenté de près de 7 milliards d’euros sur la période 2019 2024.

Ensuite, le Gouvernement a pris acte du constat d’urgence et a poursuivi la mise en place des actions complémentaires instaurées en 2023 : un soutien exceptionnel de 100 millions d’euros à destination des pour répondre aux besoins les plus urgents, mais aussi des actions pérennes pour réussir la transition démographique à venir, au travers des commissions dédiées au suivi de la situation financière des structures en difficulté installées à la fin du mois de septembre 2023 dans chaque département.

La direction générale de la cohésion sociale a également mis en place un groupe de travail associant les fédérations du secteur, des ARS et des conseils départementaux. Cinq sous groupes ont été formés, et les premières transformations sont d’ores et déjà mises en œuvre.

pour l’autonomie (CNSA) et un rapport du Gouvernement seront remis au Parlement en 2028, pour préparer sa généralisation et sa pérennisation. Les moyens de tous les Ehpad sont par ailleurs renforcés au travers de la création de 6 500 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires, conformément à l’engagement du Président de la République de créer 50 000 emplois complémentaires d’aides soignants et d’infirmiers.

Je me fais aujourd’hui le porte voix des responsables du centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle Aquitaine, région dont je suis élue, tout comme Mme Darrieussecq. Dans un contexte marqué par des restrictions budgétaires qui affectent nos concitoyens, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année à venir ne fait pas exception et subira, lui aussi, des coûts budgétaires. Le centre de dépistage, qui remplit une mission cruciale de santé publique, se trouve ainsi confronté à une forte réduction de ses moyens financiers mettant en péril l’ensemble de la chaîne de dépistage en Nouvelle Aquitaine. Ce centre est pourtant un acteur incontournable de la prévention. La Nouvelle Aquitaine s’est distinguée cette devenant la première région de France du point de vue de la progression des taux de dépistage. Le premier trimestre de 2024 a ainsi vu le dépistage du cancer du sein augmenter de 14 %, tandis que celui du cancer colorectal progressait de 50 %. Madame la ministre, alors que 40 % des cancers sont encore évitables et que tant de nos concitoyens perdent leur combat contre cette maladie en quelques mois, il est primordial d’intensifier nos efforts en matière de prévention. La stratégie décennale de lutte contre les cancers de 2021 à 2030 fixe des objectifs ambitieux : réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables et réaliser un million de dépistages supplémentaires d’ici à 2025. pourquoi réduire le budget du centre de dépistage et de prévention de Nouvelle Aquitaine, le seul en France, à ma connaissance, à être directement touché par une baisse de financement ? Vous ne devez pas faire des économies au détriment de la santé des Français ! Je demande donc au Gouvernement, madame la ministre, de reconsidérer cette décision et de permettre à ce centre de continuer de jouer son rôle essentiel dans la lutte contre le cancer.

contre le cancer, le Gouvernement avait annoncé une nouvelle organisation des dépistages organisés des cancers. Cette stratégie prévoit le transfert, à l’assurance maladie, du pilotage d’un certain nombre de missions et des crédits qui étaient alloués

Au regard de ce recentrage d’activités, l’ARS de Nouvelle Aquitaine a engagé un certain nombre d’actions pour permettre au CRCDC de Nouvelle Aquitaine de s’adapter. Aujourd’hui, ce centre se trouve effectivement dans un état déficitaire, avec un budget de 11 millions d’euros, alors que le financement délégué par l’ARS s’élève à 9 millions d’euros. Cette situation est le résultat d’un décalage important entre les orientations prises par le centre et celles qui sont prévues par l’ARS. Je fais notamment référence au transfert d’une partie de leurs missions aux ARS et à l’assurance maladie, qui devait s’accompagner d’une stabilisation des effectifs des CRCDC.

Ce sont autant d’accumulations d’actions non prévues dans le cahier des charges et pourtant mises en place par le centre qui ont conduit à ce contexte de déficit important. L’ARS de Nouvelle Aquitaine, en lien avec la direction des affaires juridiques (DAJ), ne manquera pas de se pencher sur la situation et de trouver des solutions pour rétablir un équilibre. Soyez assurée, madame la sénatrice, que le Gouvernement – en particulier Mme Darrieussecq – est pleinement engagé en faveur de la prévention et du dépistage, que nous souhaitons renforcer toujours davantage.

Pour y faire face, depuis 2024, le ministre de la santé a proposé un nouveau zonage des chirurgiens dentistes aux membres des comités d’accompagnement territorial des soins

zonage intermédiaire. Ce classement n’est pas cohérent avec les réalités vécues sur cette partie du territoire, et pour cause : la ville de La Flèche draine davantage de patients que le TVS qui la délimite, du fait qu’elle est entourée de TVS très sous dotés et que les quelques praticiens qui exercent alentour partiront prochainement à la retraite. Je veux donc porter à votre attention ce fait : dans l’hypothèse où ce nouveau zonage serait acté, il conduirait inévitablement au déménagement du seul cabinet fléchois dans le département voisin de Maine et Loire, au sein d’une nouvelle structure située en zone

au plus près de ces territoires, qui déterminent les zones éligibles à la mise en œuvre des mesures incitatives. L’objectif est, bien sûr, de favoriser une meilleure répartition des professionnels de santé, permettant ainsi un meilleur accès aux soins pour les personnes qui vivent dans des territoires sous dotés. En 2024, l’ARS des Pays de la Loire a soumis aux représentants de la profession et aux instances de démocratie sanitaire une proposition de zonage qui concerne les chirurgiens dentistes. Je rappelle qu’ils se sont appuyés sur la méthode de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL), calculé à l’échelle des territoires de vie santé (TVS). Sont prises en compte l’activité des chirurgiens dentistes, la consommation de soins de la population et la distance entre les communes. Cette méthode permet d’apprécier objectivement la réponse aux besoins des populations en fonction de l’offre de soins du territoire. Ainsi, à l’échelle nationale, la borne maximum de l’APL pour les zones « sous dotées » et « très sous dotées » s’élève à 52,19 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants. Pour 2022, l’APL du TVS de La Flèche s’élève à 53,22 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, soit un niveau supérieur à l’ensemble des TVS du département de l’Indre que vous prenez en exemple, dont le mieux doté compte 49,84 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants. Cependant, les données pour 2023 seront bientôt disponibles : elles permettront aux ARS d’actualiser leur zonage si l’évolution de l’APL le justifie. Le ministère et les services déconcentrés seront donc particulièrement attentifs

soins. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer une fois de plus l’attention du Gouvernement sur la situation préoccupante à l’hôpital Louis Constant Fleming à Saint Martin. Un contrôle de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) est réclamé par la collectivité, les partenaires sociaux et moi même depuis un certain temps, en vain. Cet établissement, le seul de l’île, est actuellement plongé dans une instabilité dangereuse. Comme il est dirigé par un second directeur par intérim, la continuité de sa gestion est compromise. L’absence de certification, le manque de projet d’établissement, l’absence d’instances telles que le comité stratégique, le comité territorial des élus et la commission médicale de groupement S’y ajoute le nombre de départ de médecins, le taux d’absentéisme, le turnover des dirigeants, les indicateurs de régression sanitaires menant au sous développement médico social et une offre de soins gravement réduite, mais aussi certains comportements qui interrogent l’éthique.

car la situation sanitaire ne cesse de se dégrader, malgré toutes les alertes et manifestations depuis 2023. La population ne veut

nombreux. L’hôpital de Saint Martin, en particulier, a bénéficié d’investissements d’ampleur ces dernières années. Au titre du Ségur, 12 millions d’euros seront mobilisés pour augmenter sa résilience et réduire les inégalités en santé. Concrètement, le plateau technique fera l’objet d’une restructuration, afin d’améliorer le traitement des urgences et des soins critiques. De même, pour mettre en conformité le service de psychiatrie, la dotation nationale du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé soit 970 000 euros – sera entièrement affectée à cet établissement d’ici à la fin de l’année. Cet investissement permettra d’améliorer significativement le fonctionnement et la sécurité globale de la psychiatrie, en respectant la dignité des patients. Alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale de l’année 2025 par le Premier ministre, soyez assurée que Mme la ministre de la santé sera particulièrement attentive à l’effectivité de ces aménagements. Pour revenir sur les dysfonctionnements que vous évoquez, il apparaît tout d’abord que, en dépit du turnover des équipes dirigeantes, l’offre de soins n’a pas été affectée. La stabilisation des équipes reste un enjeu majeur pour cet établissement, mais nous savons pouvoir compter sur les professionnels pour parvenir à des solutions pérennes. Les effectifs restent quant à eux constants depuis plusieurs années, de même que l’activité, qui se stabilise tant pour le nombre de passages aux urgences que pour les consultations. Je terminerai en évoquant l’absence de certification de la Haute Autorité de santé (HAS), qui s’explique par un manquement à certains critères impératifs. Mais ces points sont en voie de correction et n’empêchent pas l’hôpital d’afficher un score de satisfaction de 76,8 %.

Madame la ministre, vous ne répondez pas à ma question ! Les Saint Martinois comptent sur vous, ils attendent de votre part une action ferme et résolue pour mettre fin à l’instabilité qui pèse sur l’hôpital. Confrontés à une offre de soins qui se dégrade dangereusement, ils espèrent que vous saurez mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer leur droit fondamental à un accès à des soins de qualité. Il y va aussi de la confiance qu’ils placent dans l’État. Madame la ministre, votre engagement et vos décisions peuvent marquer un tournant décisif pour sortir Saint Martin de cette crise sanitaire et permettre à ses habitants de retrouver la sérénité

Depuis la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les perruques des patients ayant subi une chimiothérapie sont remboursées par la sécurité sociale, mais le montant de ce remboursement dépend de la composition de la perruque. Les perruques dites de classe 1, composées uniquement de cheveux synthétiques, dont le prix est plafonné à 350 euros, sont prises en charge intégralement. Les perruques de classe 2, qui contiennent au moins 30 % de cheveux naturels, sont remboursées à hauteur de 250 euros, mais uniquement si le prix de vente ne dépasse pas 700 euros. Dans les faits, les perruques synthétiques entièrement remboursées par la sécurité sociale sont peu choisies, car elles sont inconfortables, voire difficilement supportables au contact prolongé de la peau. de la peau. Les patientes choisissent ainsi non pas les perruques de classe 2, mais plutôt des perruques en cheveux naturels, dont le coût varie entre 1 000 euros et 3 000 euros. Comme ces perruques en cheveux entièrement naturels sont hors nomenclature, la sécurité sociale n’en rembourse rien, et nombre de patients y renoncent. Madame la ministre, il me paraîtrait équitable que tout type de perruque, quelle qu’en soit la composition, soit remboursée sur une même base.

L’accompagnement des patients ayant subi une chimiothérapie, en offrant des produits de qualité et adaptés, est essentiel. Ces accessoires sont indispensables pour le bien être des personnes malades ; ils font partie intégrante de leur parcours de soins. C’est pourquoi le Gouvernement a agi, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, en faveur de la prise en charge de ces produits. Comme vous l’indiquez, les prothèses capillaires sont aujourd’hui prises en charge par la liste des produits et prestations, avec différentes spécifications techniques : pour la classe 1, un prix limite de vente aligné sur la base de remboursement ; pour la classe 2, un reste à charge encadré. de répondre aux problématiques que vous soulevez, et ainsi favoriser l’équité d’équipement et l’accès à des soins adaptés, des travaux sur la mise en œuvre réglementaire des dispositions prévues en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) sont en cours. Leur objectif est d’améliorer les spécifications techniques des produits permettant ainsi une meilleure qualité et un meilleur confort pour les patients. Il est également de réduire le reste à charge. L’ouverture d’une prise en charge pour les perruques en cheveux naturels est ainsi prévue. Ces éléments se sont matérialisés par la publication d’un avis de projet de révision de nomenclature en septembre dernier, sur lequel la Haute Autorité de santé (HAS) rendra un avis dans les semaines à venir. Cette dernière pourra apporter des recommandations complémentaires. Les travaux pourront alors être finalisés à la suite d’une négociation tarifaire avec les acteurs du secteur et aboutir à une publication prochaine. Sachez que le ministère de la santé et ses services sont très engagés sur le sujet. Comme vous, ils seront très attentifs à l’avis qui sera rendu

La deuxième campagne nationale de vaccination scolaire contre les infections à papillomavirus humains (HPV) est en cours de déploiement dans les collèges publics et les collèges privés volontaires. La vaccination des jeunes contre le HPV est importante, car elle permet de prévenir 90 % des infections à l’origine d’un cancer au cours de la vie. Son efficacité est proche de 100 % lorsqu’elle est réalisée avant le début de la vie sexuelle. Elle est organisée au sein même de l’établissement scolaire et proposée aux élèves de cinquième lorsque leurs parents y ont consenti. soit en progression, la précédente campagne vaccinale n’a pas atteint son objectif, à savoir vacciner 30 % des 800 000 élèves de cinquième. En effet, votre prédécesseur a annoncé, en mars 2024, que 117 000 élèves, c’est à dire 15 % de la cible, étaient vaccinés. Par ailleurs, cette première campagne a mis en évidence des disparités importantes. Les

Dans le département des Hauts de Seine, des différences significatives sont constatées d’une commune à l’autre. Malgré les efforts déployés par les équipes éducatives, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les services départementaux de médecine scolaire, des difficultés persistent. Madame la ministre, pouvez vous nous indiquer si les freins expliquant les résultats décevants de cette première campagne vaccinale ont été identifiés ? Et quelles mesures sont elles prévues pour améliorer l’information et la couverture vaccinale des collégiens sur l’ensemble du territoire, en particulier

Comme vous le soulignez, la vaccination contre le papillomavirus couvre 90 % des infections à l’origine de cancers ; c’est une vaccination sûre, les données produites par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) le montrent. C’est dans ce cadre que la première campagne de vaccination contre les HPV dans les collèges publics et privés volontaires a été lancée pendant l’année scolaire 2023 2024.

Cette campagne a aussi permis d’évoquer les risques de cancers liés aux HPV et d’informer les jeunes, ainsi que leurs parents, sur l’importance d’être vacciné jeune, avant toute exposition aux HPV. Elle a entraîné une forte dynamique de vaccination en ville, avec une hausse de 20 % en 2023 par rapport à 2022. Au total, plus de 400 000 adolescents, âgés de 12 ans en 2023, ont reçu au moins une dose de vaccin représentant 48 % de cette tranche d’âge – soit une augmentation considérable de 17 points de la couverture vaccinale. Vous avez raison, nous avons encore des efforts à fournir pour atteindre notre objectif de vacciner 80 d’une tranche d’âge d’ici à 2030, afin d’éradiquer les cancers liés aux HPV. C’est pourquoi une nouvelle campagne de vaccination des élèves de cinquième a été lancée lors de la rentrée scolaire 2024 2025 dans les collèges.

– séances d’information et de sensibilisation des élèves de sixième, envoi d’un courrier d’information aux parents dès le mois de juin… Cette nouvelle campagne représente l’occasion d’aller vers les populations insuffisamment vaccinées en leur offrant une vaccination gratuite, gratuite, sûre et efficace. Nous y consacrerons les moyens nécessaires. Sachez, madame la sénatrice, que le ministère de la santé et ses services sont tout à fait mobilisés sur ce sujet. La parole

rapide et profonde de leurs comptes. En 2023, quelque 92 % d’entre eux, tous statuts confondus, prévoyaient une fin d’année en déficit. Les conséquences de cette situation sont particulièrement inquiétantes en termes de recrutement, de valorisation du personnel, de tension de trésorerie ou d’investissement dans de nouveaux bâtiments, si nécessaires pourtant pour la mise en conformité et le bien être des résidents. Alors même que tous les rapports parus ces derniers mois convergent pour confirmer l’impératif absolu d’investir pour le grand âge, en identifiant de nouvelles sources de financement, afin notamment de créer 100 000 emplois d’ici à 2030, force est de reconnaître Si, en 2023, un fonds d’urgence de 100 millions d’euros a été créé, ce dernier a servi à soutenir les Ehpad dans les situations les plus critiques. Dans le département de la Mayenne, plusieurs structures relevant de

Les Ehpad ont notamment bénéficié d’un plan d’aide exceptionnel dans le cadre du Ségur de la santé entre 2021 et 2024. Le volet médico social s’est élevé à 1,5 milliard d’euros.

Les élus sont tenus informés des travaux – examen des difficultés de trésorerie et souplesses accordées dans le paiement des dettes sociales ou fiscales. Ces commissions ont été pérennisées en janvier 2024. Elles feront également l’objet d’un suivi réalisé au niveau national par une cellule ministérielle. La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a également mis en place un groupe de travail associant les fédérations du secteur, les ARS et les conseils départementaux. Cinq sous groupes ont été formés ; les premières transformations sont d’ores et déjà mises en œuvre.

Les moyens de tous les Ehpad sont par ailleurs renforcés au travers de la création de 6 500 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires, conformément à l’engagement du Président de la République de créer 50 000 emplois complémentaires d’aides soignants et d’infirmiers.

L’ensemble de ces dispositions vise à donner de la stabilité à une activité indispensable à l’enseignement en faveur des jeunes en situation de handicap. Hélas ! les décrets et circulaires qui devraient découler de nos débats et décisions parlementaires

d’autre part, par les rectorats, qui sont l’instance d’appartenance de la catégorie professionnelle, ainsi que par les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), qui sont chargés de l’organisation fonctionnelle de la répartition du travail.

Pouvez vous nous garantir, madame la ministre, que le Gouvernement ira dans cette direction et prendra les mesures pour garantir cette meilleure stabilité des AESH que tout le monde appelle de ses vœux ? La parole est à Mme la ministre déléguée.

Aujourd’hui, 513 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, un chiffre en constante augmentation depuis 2017. Parmi eux, 336 732 bénéficient d’une notification de la MDPH, soit 65 % des élèves en situation de handicap. Les AESH sont des professionnels essentiels à la réussite des élèves en situation de handicap. À la fin de l’année 2024, ce sont 140 000 AESH qui accompagneront quotidiennement les élèves pour les aider à gagner en autonomie dans leurs apprentissages. Entre 2022 et 2025, quelque 13 000 emplois auront été créés pour répondre aux besoins d’accompagnement sans cesse croissants des élèves en situation de handicap. La dynamique se poursuit en 2025, avec la création de 2 000 La gestion administrative des AESH a été progressivement confiée aux rectorats dans le cadre d’un service académique dédié, affirmant ainsi la pleine reconnaissance de ces personnels au sein de l’éducation nationale, au même titre que les enseignants. Cela s’est accompagné d’une évolution de leur statut avec la CDIsation de ces personnels dès trois ans d’activité professionnelle depuis la rentrée 2023, ainsi que d’une revalorisation statutaire et financière, afin de stabiliser le cadre d’emploi et de fidéliser ces personnels. Le ministère de l’éducation nationale est tenu de mettre en œuvre ces notifications dès qu’elles sont portées à sa connaissance. Afin de garantir une réponse au plus près des besoins de chaque élève, l’emploi du temps des AESH est alors organisé en conséquence au sein des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), ou, depuis la rentrée 2024, dans quatre départements préfigurateurs au sein des pôles d’appui à la scolarité Cette nouvelle organisation en PAS permet une meilleure réactivité dans l’accompagnement des élèves, ainsi qu’une réponse rapide de première intention ou à plus long terme.

et de la petite enfance. Madame la ministre, mes chers collègues, à compter du 1 janvier 2025, la loi n° 2023 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confie la compétence « petite enfance » aux communes. Celles ci deviendront ainsi les « autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant ». Or, selon les configurations territoriales, cette compétence a pu être précédemment confiée à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), afin de garantir un accès diversifié et équitable aux habitants d’un même territoire. Dès lors, qu’en sera t il pour ces EPCI ? Pourront ils assurer la continuité du service public en poursuivant l’exercice de cette compétence ? ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Madame la ministre, quels seront les moyens alloués à cette réforme ?

et la création de 35 000 places en établissement d’accueil du jeune enfant d’ici à 2027. On est malheureusement bien loin du compte ! Les élus que nous sommes connaissent tout particulièrement la réalité d’une telle compétence. Nous n’avons pas attendu votre loi pour créer des places d’accueil pour nos enfants. Si le nombre de places d’accueil pour les jeunes enfants est encore aujourd’hui insuffisant, ce n’est clairement pas un manque d’intérêt des élus pour la petite enfance, bien au contraire ! C’est avant tout une question de moyens financiers et humains. J’aurais donc deux questions, madame la ministre. Quel accompagnement de ces objectifs prévoyez vous dans la durée ? Et quels moyens seront dédiés aux communes, de manière pluriannuelle, pour le fonctionnement d’une telle ambition ? La parole

Par exemple, sur votre territoire du Val d’Oise, on compte 41 places d’accueil pour 100 enfants de moins de trois ans. Les dépenses de la branche famille ne diminuent donc pas entre 2024 et 2025, ce qui souligne l’importance que le Premier ministre porte à ces politiques publiques. En fonction du nombre d’habitants, une commune doit obligatoirement exercer tout ou partie de quatre compétences : recenser les besoins ; informer et accompagner les familles ; planifier le développement des modes d’accueil ; enfin, soutenir la qualité de ces modes d’accueil. La concrétisation du service public de la petite enfance en 2025 sera rendue possible grâce à l’engagement des communes, ou des intercommunalités le cas échéant, dans le cadre de leurs nouvelles compétences d’autorités organisatrices. Le Gouvernement a précisé, sur une foire aux questions, les modalités de mise en œuvre de la compétence, afin de répondre aux principales questions que les communes et intercommunalités peuvent se poser.

à partir desquels la répartition de cet accompagnement financier sera réalisée. Les critères envisagés sont le nombre de naissances et le potentiel financier des communes, afin d’orienter davantage l’accompagnement financier de l’État vers les communes disposant des ressources les moins élevées.

que, dans un délai de vingt ans, 100 000 nouvelles victimes de l’amiante pourraient être identifiées. En effet, si l’amiante est interdit depuis vingt sept ans maintenant, le nombre de ses victimes s’accroît sans cesse,… C’est vrai ! … d’une part, car les maladies peuvent se déclarer plusieurs décennies après l’exposition, et, d’autre part, car 20 millions de tonnes d’amiante seraient encore présentes dans les bâtiments.

revenait sur une victoire obtenue par l’Andeva, c’est désormais l’article 24 du PLFSS 2025 qui concentre toute notre attention. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de faute inexcusable de l’employeur sous forme de rente risquerait,

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Fagnen, l’attention de la ministre du travail et de l’emploi est attirée sur la prévention des expositions professionnelles à l’amiante et sur la réparation de ces expositions. Un décret du 4 mai 2012 a relevé significativement le niveau de prévention en matière d’exposition des travailleurs à l’amiante. Il a abaissé la valeur limite d’exposition professionnelle à 10 fibres d’amiante par litre d’air sur huit heures et a imposé une méthode d’analyse capable de décompter toutes les fibres d’amiante cancérigènes. L’inspection du travail contrôle attentivement le respect de cette réglementation, avec près de 11 000 interventions en 2022. La cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Caata) est un dispositif de réparation à titre collectif, justifié par des expositions à l’amiante importantes intervenues Ce dispositif s’applique, à titre individuel, aux salariés atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante et, à titre collectif, aux salariés des établissements inscrits sur les listes fixées par les arrêtés du 3 juillet 2000 et 7 juillet 2000 et régulièrement mises à jour. Les salariés exposés à l’amiante peuvent, depuis 2010, demander la réparation du préjudice d’anxiété, quand les ouvriers de l’État Caata vaut reconnaissance d’un lien établi entre l’exposition à l’amiante et la baisse de l’espérance de vie, ce qui permet d’être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété.

En revanche, des sites relevant historiquement de DCNS sont inscrits, depuis 2001, dans l’arrêté ouvrant droit au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité Les partenaires sociaux ont réaffirmé, en mai 2023, puis en 2024, leur attachement au caractère dual de l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 retranscrit fidèlement leur accord. La parole

concerne la formation. La certification Qualiopi est obligatoire pour tous les prestataires proposant une formation de développement de compétences. Elle leur permet d’être éligibles aux financements publics. Depuis son entrée en vigueur, en 2021, ce dispositif a été révisé à neuf reprises, entraînant de nombreuses superpositions de formalités et de contraintes. La certification impose la validation de 32 indicateurs et de multiples points de contrôle, avec de nombreuses redondances. Si l’instauration d’un cadre rigoureux est nécessaire, nous constatons aujourd’hui plusieurs écueils regrettables,

temps plein (ETP) administratif pour 56 apprenants en 2014, contre 5,5 pour 150 élèves aujourd’hui. Si l’intention initiale était d’assainir le secteur des centres de formation, c’est véritablement un échec Des structures spécialisées dans l’accompagnement pour l’obtention de la certification Qualiopi prolifèrent, créant un véritable marché parallèle ; des centres proposent parfois des formations en 100 % à distance, lesquelles peuvent être mal ou peu dispensées ; des élèves insuffisamment formés ne valident pas pas leurs examens… Pourtant, les centres concernés disposent du même niveau de soutien de l’État ! On peut donc légitimement s’interroger sur l’efficience de ces dépenses. Madame la ministre, comment le Gouvernement imagine t il faire évoluer le dispositif Qualiopi pour garantir sa performance ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Billon, depuis son entrée en vigueur au 1 janvier 2022, les prestataires d’actions concourant au développement des compétences doivent obtenir la certification qualité Qualiopi pour accéder aux fonds publics et mutualisés gérés par les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316 1 du code du travail. Je tiens à souligner que les critères et indicateurs sont restés stables ; le référentiel est toujours le même. Seul le guide de lecture a évolué, de manière à être plus lisible et précis en fonction des demandes des acteurs de la formation. Il semble également important de préciser que l’augmentation du nombre d’organismes de formation est surtout liée à l’obligation, pour les sous traitants, de se déclarer. Par ailleurs, tous ne demandent pas la certification sur les 125 000 organismes actifs recensés en octobre 2024, seuls 44 633 sont certifiés Qualiopi. Selon une étude du Centre d’études et de 2023, seuls 6,5 % des organismes de formation ont recruté durablement une personne dans le cadre de la certification. Le sujet de la qualité est une préoccupation majeure de Mme la ministre du travail et de l’emploi, qui entend poursuivre les travaux engagés en lien avec les partenaires sociaux et les représentants des financeurs ainsi que de l’offre de formation. La question de la qualité de l’accompagnement des apprentis, le respect des 14 missions assurées par les centres de formation d’apprentis (CFA) et l’adéquation des moyens mis en œuvre au regard des certifications proposées constituent des priorités. Plus largement, une meilleure coordination des contrôles et des audits conduits en matière de formation est également un axe de travail. La parole

L’enseignement privé est aujourd’hui financé à plus de 76 % par des fonds publics. Pourtant, il est difficile d’avoir des données claires sur les moyens alloués et les effectifs réels, ainsi que sur le nombre de classes et d’enseignants qu’il représente, en particulier Je ne suis pas la seule à le déplorer : je rappelle ici que la Cour des comptes elle même, dans son désormais fameux rapport sur l’enseignement privé de 2023, estimait que les inégalités entre enseignement public et privé ne cessaient de s’accroître, fondées sur une répartition des moyens

très importants entre les collèges publics et les collèges privés sous contrat, les dotations semblent quasi identiques. Les lycées généraux et technologiques publics seraient également les grands perdants. Si la méthode de calcul utilisée pour définir les moyens des établissements privés s’appliquait aux établissements publics, ces derniers auraient droit à la création de 12 850 postes d’enseignants. À l’inverse, si le privé était soumis à la même règle, ce sont 2 040 de ses postes qui devraient être supprimés. À Paris, à la rentrée, dans l’enseignement public, on a compté 127 classes en moins dans le premier degré. Dans le même temps, l’enseignement privé parisien a connu un déconventionnement d’une cinquantaine de classes seulement. Il est temps de mettre fin à ce déséquilibre intolérable entre public et privé, qui conduit de fait à faire absorber la baisse démographique quasi exclusivement par l’enseignement public. Parce que la démographie ne peut tout justifier,

Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Brossel, comme vous le savez, la répartition des moyens entre les enseignements public et privé est inchangée au niveau national : elle répond au principe de parité

concerne plus spécifiquement l’enseignement privé dans l’académie de Paris, qui est marquée par une forte proximité géographique entre établissements privés sous contrat et établissements publics, un travail de convergence avec le schéma d’emplois prévu dans l’enseignement public a été mené, afin d’aboutir, pour la rentrée scolaire 2024, au retrait de 50 équivalents temps plein (ETP). Durant l’année scolaire 2023 2024, le taux d’encadrement dans le premier degré de l’enseignement privé était de 25,5 élèves par classe, soit près de 6 élèves de plus par classe que dans l’enseignement public. Dans le second degré, les taux d’encadrement sont très nettement favorables à l’enseignement public au collège. Au lycée, en revanche, le nombre d’élèves par classe est moins important dans l’enseignement privé. Par ailleurs, et même si la composition sociale des établissements publics parisiens est déjà très favorisée, avec un indice de position sociale (IPS) moyen au collège de 117,2, contre 100,8 au niveau national, on constate un écart important avec les établissements privés, dont l’IPS moyen au collège est de 147,5. Dans ce contexte, le ministère de l’éducation nationale veillera, dans le cadre des travaux de préparation de la prochaine rentrée scolaire, à maintenir un équilibre entre les deux secteurs d’enseignement et à œuvrer en faveur d’une amélioration de la mixité sociale et scolaire dans cette académie. La parole

l’enquête judiciaire pour abus de confiance aggravé et blanchiment se poursuit, soit l’OQTF doit être appliquée ! En toute hypothèse, nous avons, depuis le 9 avril 2024, une convention d’entraide avec le Kazakhstan.

à l’encontre de ce ressortissant kazakhstanais, fait suite au refus d’extrader ce dernier opposé par l’autorité judiciaire française, refus qui a été suivi d’une dénonciation officielle des faits par les autorités kazakhstanaises. L’ouverture d’une telle procédure judiciaire, toujours en cours et couverte par le secret de l’instruction, est l’illustration flagrante de l’exacte application qui a été faite par la France du principe « extrader ou juger », prévu par l’article 113 8 2 du code pénal. Si les demandes d’extradition entre la France et le Kazakhstan ne disposent toujours pas de fondement conventionnel dédié, il n’en va plus de même des demandes d’entraide pénale internationale, qui peuvent dorénavant être transmises sur la base de la convention bilatérale d’entraide signée entre nos deux pays le 28 octobre 2021 et qui est entrée en vigueur le 1 septembre 2024. Celle ci ne pourra que faciliter et fluidifier la coopération franco kazakhstanaise en matière d’entraide aux fins d’enquête, éventuellement dans le cadre de l’information judiciaire évoquée. concerne, enfin, la question de la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français délivrée à l’encontre de ce ressortissant kazakhstanais, le ministère de la justice n’est pas compétent pour y répondre, s’agissant d’une procédure administrative. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question s’adressait au ministre de la justice, garde des sceaux. Elle porte sur la sécurisation de nos prisons, en particulier sur les livraisons par drone. En effet, ces engins volants commandés à distance sont de plus en plus utilisés par des réseaux de délinquants pour faire parvenir aux détenus toutes sortes de marchandises illicites : armes, téléphones, drogue… Force est de constater que nos prisons sont constamment en proie à d’innombrables trafics et exactions, qui ne doivent plus durer. À titre d’exemple, dans le département de la Meuse, le centre de détention de Saint Mihiel recense, depuis le 1 janvier dernier, au minimum 26 livraisons interceptées par le personnel pénitentiaire. Cela en fait, à l’échelle du Grand Est, un établissement particulièrement affecté par ce phénomène. Cette situation suscite de fortes inquiétudes chez des agents pénitentiaires, qui doivent aussi faire face à une violence croissante, laquelle se manifeste tant à l’encontre des surveillants que des détenus eux mêmes. des livraisons par drone, mais aussi face au développement de trafics, des moyens technologiques et techniques existent et ont été déployés, tels que les filets au dessus des bâtiments, les fusils permettant de neutraliser les aéronefs ou encore les brouilleurs de drones et de portables. Ces dispositifs constituent des outils efficaces pour lutter contre les trafics et améliorer la sécurité de nos agents. Certains établissements en sont d’ores et déjà dotés, mais ils doivent être généralisés. Madame la ministre, nous ne pouvons laisser nos prisons gangrenées par les trafics. Certaines d’entre elles deviennent même les lieux d’où sont pilotés et commandités des actes de grand banditisme, comme à Marseille dernièrement. Envisagez vous la systématisation des moyens pour neutraliser les drones au sein des établissements pénitentiaires ? Si oui, selon Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Menonville, mon collègue garde des sceaux tient à vous remercier de votre question, qui lui permet d’affirmer devant cet hémicycle son profond attachement à la protection des personnels et des établissements pénitentiaires contre toute forme d’acte malveillant, ainsi qu’à la lutte contre la poursuite de toute activité criminelle contre la poursuite de toute activité criminelle ou délictuelle depuis la détention. La lutte contre la livraison par drone est une priorité. Si les fusils neutralisants sont des outils utilisés par les services de la police et de la gendarmerie nationales contre ces aéronefs, leur usage n’est pas adapté à l’administration pénitentiaire. Le délai d’intervention pour les agents est trop court – moins de dix secondes. Le déploiement d’autres technologies a donc été privilégié. À ce jour, 47 sites sont équipés d’un système anti drones pour faire face au survol des bâtiments et endiguer cette menace par la neutralisation de la trajectoire des appareils. Un plan volontariste de déploiement de dispositifs anti drones est en cours pour équiper des établissements particulièrement ciblés par ce problème. Dans ce cadre, le centre de détention de Saint Mihiel a été identifié et sera équipé, au cours de l’année 2025, d’un dispositif de caractérisation et de neutralisation des drones. Le centre de détention de Montmédy est quant à lui doté d’un dispositif de détection et de neutralisation des communications illicites, utile pour les brouillages de téléphones. Des travaux importants commencés en 2023 et achevés en 2024 ont également permis la pose de filets anti projections. S’y ajoutent, enfin, des opérations de fouille de cellules et de secteurs de détention réalisées par les agents, destinées à la saisie des objets ou substances illicites. La parole

mer. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. le ministre des outre mer. Monsieur le ministre, je souhaite relayer avec force les appels à l’aide des communes calédoniennes. Le 5 août dernier, les deux associations de maires de Nouvelle Calédonie, qui rassemblent les 33 communes du territoire, ont alerté le Gouvernement sur l’extrême fragilisation des budgets des communes à la suite des émeutes du 13 mai et ont formulé plusieurs demandes de soutien financier. Parmi elles figure une demande d’augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour le projet de loi de finances 2025, afin de compenser les pertes de recettes liées à la division par deux de la part versée par la Nouvelle Calédonie, dont les recettes fiscales se sont effondrées du fait de la destruction de 25 % du tissu économique. Ce sont ainsi 25 % des recettes des communes qui font défaut pour finir le budget en cours ! Les maires vous l’ont d’ailleurs rappelé lors de votre visite. Le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a également appuyé auprès de l’État une demande d’aide exceptionnelle de 34 millions d’euros pour le budget en cours des communes du territoire. Vous avez annoncé un engagement massif de l’État aux côtés des communes calédoniennes en matière d’investissement, avec notamment la prise en charge à 100 % de la remise en état du bâti scolaire, et à 70 % de celle des autres bâtiments publics, après la mobilisation des contrats d’assurance. Monsieur le ministre, ma question sera double. Comment comptez vous soutenir financièrement le budget de fonctionnement des communes calédoniennes pour la fin de l’année 2024 ? compte tenu des montants de DGF, qui restent stables dans le PLF pour 2025, comment allez vous soutenir leur fonctionnement pour l’année 2025, sachant que ces collectivités sont l’échelon essentiel du vivre ensemble et constituent le point d’appui de la reconstruction de la Nouvelle Calédonie Les communes de Nouvelle Calédonie comptent sur vous

À cette occasion, j’ai voulu rassurer les communes, en leur confirmant que le soutien de l’État, dans le cadre d’un accompagnement spécifique, sera mis en place. Les conditions de ce soutien s’inspirent quelque peu de ce qui s’est passé dans l’Hexagone au mois de juin 2023, après les événements liés au décès du jeune Nahel Merzouk. les communes bénéficieront d’une aide permettant de contribuer à la remise en état et/ou, selon les circonstances, à la reconstruction des bâtiments publics détruits et endommagés, conformément d’ailleurs à la note d’instruction que j’ai signée le 17 octobre dernier depuis Nouméa. J’ai J’ai évidemment demandé à notre Haut Commissaire de faciliter autant que possible le traitement des demandes de subventions, par la mise en place d’un guichet unique destiné à centraliser le recensement des besoins et à accompagner les collectivités concernées. Ce guichet leur permettra d’accéder aux informations et dispositifs utiles

pour procéder à l’évaluation du montant des dégâts et accompagner les collectivités dans la durée. J’ajoute une petite précision : les dégâts ont conduit à une baisse de 15 % du produit intérieur brut de la Nouvelle Calédonie… Il faut avoir ce chiffre en tête. Les collectivités devront en tout état de cause mobiliser en premier lieu les contrats d’assurance souscrits pour se couvrir contre les dommages. Nous savons bien qu’il y a des difficultés avec les assureurs : nous sommes en train de nous en occuper. Pour ce qui concerne les établissements scolaires, l’État financera intégralement et sans limite limite le reste à charge des collectivités après l’intervention des assurances. Pour les autres biens et équipements, le taux de subventions accordées par l’État sera modulé en tenant compte évidemment des crédits budgétaires disponibles, du caractère structurant des infrastructures concernées, de leur état de vétusté de la situation financière des collectivités maîtres d’ouvrage. Il pourra, à titre exceptionnel, être porté à 100 % de l’assiette de dépenses subventionnables. Dans ce cadre, les communes et leurs groupements ont jusqu’au 17 novembre pour adresser au haut commissariat les demandes de subventions. Ce délai est suffisant, mais il est assez court… Il ne faut pas mollir. Au titre de la solidarité nationale et de l’urgence, cet accompagnement s’inscrit dans un plan global de soutien de l’État. Je rappelle que, jusqu’au mois de septembre dernier, l’État s’était engagé à la hauteur de 400 millions d’euros, qu’un

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le ministre, chaque semaine, des dizaines, voire des centaines de personnes, fuyant la misère ou l’oppression, après un périple dangereux à travers l’Afrique et l’Europe, de traverser la Manche, au péril de leur vie, pour rejoindre la Grande Bretagne dans l’espoir d’une vie meilleure.

Le 8 octobre dernier, à la suite de quatre nouvelles disparitions, dont celle de deux enfants, les maires du littoral ont exprimé leur sentiment d’abandon et leur colère et demandé à l’État d’agir. Ma question est simple, monsieur le ministre : que leur répondez vous ? Quels moyens allez vous déployer pour éviter ces drames, lutter efficacement contre les passeurs et protéger les migrants ? La parole

Depuis l’accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume Uni, il n’y a pas de cadre juridique européen. Il en faudra un, et nous défendons le principe de la nécessité d’un partenariat migratoire entre l’Union européenne et le Royaume Uni.

Les habitants, ainsi que les élus locaux, sont exaspérés. Depuis près de trente ans, les municipalités successives demandent un commissariat de plein exercice. La mairie a consenti des efforts financiers depuis 2018 pour se doter d’une police municipale, mais cette dernière n’a pas vocation à se à se substituer aux missions de la police nationale. Accéder à cette revendication serait un symbole fort, démontrant que l’État n’abandonne pas ces quartiers.

le territoire. Le commissariat de Sevran est aujourd’hui sous l’autorité de celui d’Aulnay sous Bois, en cours de reconstruction. Les effectifs actuels de soixante policiers affichés à Sevran sont donc contextuels

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, je vous demande d’écouter la demande incessante des acteurs de terrain et d’instaurer un commissariat de plein exercice à Sevran. La parole est

en vue du démantèlement des trafics qui ont conduit à ces violences. Je veux saluer, à mon tour, les polices municipales de Sevran et d’Aulnay sous Bois, qui travaillent main dans la main avec la police nationale dans le cadre de la sécurisation des établissements scolaires. Nous sommes prêts, madame la sénatrice, à aller plus

à la sauvette à Paris. Installés à proximité des zones touristiques, comme la butte Montmartre, la tour Eiffel ou encore sur les ponts parisiens, ces marchands illégaux vendent des denrées alimentaires, des articles de souvenirs, des produits qui sont très souvent de contrefaçon ou de très mauvaise qualité. Les boutiques de souvenirs, les commerçants et les restaurateurs qui, eux, bénéficient d’une autorisation d’occupation s’inquiètent très légitimement d’une concurrence déloyale de plus en plus forte.

plus anxiogène. Quelle image de Paris et de la France donnons nous au reste du monde ? Monsieur le secrétaire d’État, quels moyens le Gouvernement entend il déployer pour lutter plus efficacement contre les vendeurs à la sauvette à Paris ?

Privés d’accès au fichier des véhicules assurés (FVA) par une décision du Conseil constitutionnel de 2021, les policiers municipaux sont dépendants des services de l’État pour obtenir ces informations. Lorsqu’ils contactent le commissariat ou la gendarmerie, la réponse n’est pas toujours immédiate, ni même garantie. Elle dépend bien évidemment de l’activité et de la charge de travail du moment, ce qui nuit nécessairement à l’efficacité de leur intervention. Monsieur le secrétaire d’État, notre mission de fabrique de la loi consiste à rendre opérable la loi sur le terrain. Je vais donc prendre deux exemples concrets.

par exemple, les policiers municipaux ne reçoivent que des informations limitées, les mêmes que celles qui sont accessibles aux garages automobiles. Les polices municipales et les maires qui les supervisent jouent un rôle essentiel dans le continuum de sécurité. Pour être pleinement efficaces, ils ont besoin de moyens adaptés. Simplifier les démarches, oui évidemment ; mais alors, pour toutes nos forces de l’ordre en vue d’une meilleure efficacité opérationnelle Monsieur le secrétaire d’État, dans un contexte où le besoin d’ordre et de respect des règles élémentaires est grandissant, où les maires sont des acteurs majeurs de la sécurité du quotidien et assurent des fonctions régaliennes, quelle mesure concrète envisagez vous de prendre pour remédier à ces lacunes et faciliter l’accès des polices municipales aux fichiers nécessaires à leur mission ?

à ce continuum de sécurité, cette chaîne au sein de laquelle les forces de police municipale jouent un rôle important. C’est pourquoi le ministre de l’intérieur a demandé à Nicolas Daragon, ministre délégué chargé

Selon la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), 19 % des étudiants ne mangent pas à leur faim ; parmi les boursiers, ce chiffre monte à 28

Où en est l’engagement du Gouvernement concernant la construction de nouveaux logements étudiants à prix accessible ? Allez vous enfin mettre en place des mesures correctives pour enrayer la dégradation des conditions de vie des étudiants ? Les jeunes sont l’avenir de notre pays

sur les effets désastreux induits par la redéfinition de la géographie prioritaire de la ruralité. La réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR) a soulevé de nombreuses contestations dans les territoires en raison de son caractère inéquitable. Depuis 2019, la commission que je préside est force d’initiative et a versé à la réflexion collective des préconisations clés en main afin d’appréhender équitablement les singularités des communes rurales. Jamais l’exécutif n’a sérieusement envisagé la recommandation consistant à rebâtir un zonage à la maille non plus intercommunale, mais communale. Les effets de bord que nous avions signalés sont apparus. Il est temps désormais d’écouter le bon sens sénatorial. En juin dernier, environ 2 200 communes ont été « rattrapées » par l’ancien Premier ministre. Cette évolution, certes nécessaire, suscité de grandes inquiétudes : en l’absence de cadre juridique adéquat, ces communes ne respectent pas les nouveaux critères de classement. Si l’on considère attentivement les deux arrêtés parus le 29 juin dernier, on constate que les communes rattrapées sont en réalité réintégrées dans le dispositif des ZRR et non dans le les place dans une situation de grande précarité juridique en l’absence de base légale. Cette aberration juridique n’est cependant pas l’unique malfaçon de cette réforme. Pour les communes concernées, la situation peut être grave et préjudiciable. Il semblerait que certaines directions régionales des finances publiques (DRFiP) refusent d’appliquer à ces communes les abattements et mesures fiscales qui découlent du classement. Cette incertitude est délétère et doit impérativement cesser. L’autorité de la parole de l’État est en jeu. Ma question est donc simple : que comptez vous mettre en œuvre pour pallier les effets pervers de cette réforme ? Quel sort réservez vous aux communes rattrapées ? Enfin, envisagez vous de garantir la sécurité juridique desdites communes en apportant les correctifs structurels nécessaires ? La parole est à M. le ministre

et a conduit à l’entrée en vigueur d’un nouveau zonage, France Ruralité et Revitalisation, au 1 juillet 2024. Près de 17 700 communes ont intégré ce zonage, qui permet aux entreprises implantées localement de bénéficier d’exonérations sociales et fiscales renforcées, afin de soutenir l’attractivité et le développement économique des collectivités rurales. Le Premier ministre a annoncé le 4 juin dernier que les 2 200 communes situées en ZRR qui n’étaient pas éligibles au nouveau zonage FRR au 1 juillet 2024 seraient maintenues dans le dispositif. Cette mesure permet d’assurer une continuité dans le soutien apporté par l’État aux politiques structurelles de développement économique et territorial en ruralité, et je veux vous assurer de la détermination de Catherine Vautrin à la faire appliquer.

j’ai conscience de l’exaspération que peut susciter la multiplicité d’antennes dans certaines zones de nos territoires. Les politiques mises en place, comme le New Deal mobile, constituent des réponses à un manque de couverture criant pour nos concitoyens.

De plus, c’est la concurrence par les infrastructures qui permet aux opérateurs de se différencier en matière de qualité de couverture, et donc de qualité de service. Dans le cadre du New Deal mobile et du dispositif de couverture ciblée, les opérateurs ont l’obligation de mutualiser leurs pylônes et installations actives lorsqu’ils sont quatre sur la zone. Par ailleurs, l’arrivée des favorise la mutualisation puisque, dans un souci de rentabilité de leur modèle financier, elles ont intérêt à avoir le maximum d’opérateurs sur leurs antennes. D’autres obligations légales sont déjà en application, comme l’obligation en zone de montagne, ou dans le cadre du déploiement 5G en zone peu dense. De plus, avant toute implantation d’antenne, un temps de dialogue est instauré la communication des dossiers d’information aux maires. Je le redis, rien n’est fait à l’encontre des décisions du maire et sans concertation locale. grâce à l’ensemble de ces mesures, 70 % des antennes sont mutualisées. Par ailleurs, 1 million de personnes supplémentaires disposent d’une couverture 4G depuis 2018. Nous continuons nos efforts pour garantir une couverture de l’ensemble de nos concitoyens. Dans l’Aisne, soixante sites ont été identifiés depuis la mise en place du dispositif sont déjà mis en service. Les opérateurs de télécommunication se sont également engagés à couvrir les axes routiers prioritaires et ferroviaires et à assurer une couverture nécessaire à l’intérieur des bâtiments. La généralisation d’une très bonne couverture 4G demeure un engagement fort

de la décentralisation. Monsieur le ministre, j’ai une proposition concrète à vous faire dans le cadre du nouveau contrat de responsabilité que le Gouvernement souhaite bâtir avec les collectivités. Sans rien coûter à l’État, elle renforcerait la confiance vis à vis des élus locaux

Ces 152 dossiers concernent des projets de communes petites et moyennes, souvent rurales, qui ne peuvent voir le jour qu’en cumulant la DETR avec une subvention départementale ou régionale. Bien sûr, le préfet a fourni le détail de ces 152 dossiers, mais une information aux élus n’est pas un avis des élus. Élargir la saisine pour avis de la commission DETR à l’ensemble des dossiers présentés serait un élément de simplification et de transparence. Le ministère de l’intérieur doit aussi veiller à notifier aux préfets le montant officiel de leur DETR avant fin mars. Par prudence, les préfets l’attendent pour faire les notifications aux maires, ce qui permettrait le lancement des travaux avant l’été.

croit également à la déconcentration et au rôle des préfets au plus proche des réalités du terrain pour soutenir les projets des collectivités. Les contreparties de l’utilisation de ces fonds du budget de l’État sont bien entendu la transparence et l’égalité de traitement

Le préfet publie ensuite en la liste des projets retenus, ainsi qu’un rapport annuel d’exécution. Cette liste permet aux membres de la commission d’être parfaitement informés. informés. Depuis la loi de finances pour 2024, les préfets doivent enfin porter à la connaissance de la commission la liste des opérations non retenues, mais dont le dossier a été déclaré complet et recevable. La commission départementale des élus est donc informée de l’intégralité des projets pour lesquels une demande de DETR a été déposée.

d’attribution de la DSIL, et que le préfet de région communique à cette commission, ainsi qu’à l’ensemble des parlementaires du département, la liste des projets subventionnés au titre de la DSIL ainsi qu’un bilan d’exécution de la dotation.

Le potentiel de cet aérodrome est toutefois bien plus important, au regard à la fois du foncier disponible – plus de 100 hectares d’un seul tenant –, de sa piste d’une longueur de 1 975 mètres, soit l’une des plus grandes de France, de sa tour de contrôle moderne, qui a du reste coûté très cher aux contribuables, et de sa

de l’échangeur autoroutier de l’A5, régulièrement engorgé aux heures de pointe. Monsieur le ministre, pouvez vous me confirmer que les intentions de l’État vont dans ce sens et que votre gouvernement s’engagera à faire de l’aérodrome de Melun Villaroche un modèle de réindustrialisation, mais aussi une infrastructure digne de la première région d’Europe ?

et de développement de l’aérodrome relève de la compétence des collectivités propriétaires du terrain. Si l’État n’a pas vocation à participer au financement d’une partie des investissements de cet aérodrome, il veille à accompagner les projets conduits par le syndicat mixte.

Plus récemment, en 2021, les services de la DGAC ont accompagné l’exploitant de l’aérodrome et les collectivités locales dans le cadre du projet partenarial d’aménagement de la zone dite Paris Villaroche, en proposant des solutions visant à optimiser l’usage du foncier disponible pour le développement économique tout en préservant les infrastructures aéronautiques.

sûreté. Les montants perçus au titre des péréquations de 2022 et 2023 s’élèvent respectivement à 277 000 euros et à 380 000 euros. La direction générale des douanes et droits indirects et la police aux frontières sont les services de l’État

La commune de Saint Saulve, située sur le territoire de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, qui a profité avant les années 2000 de nombreuses implantations industrielles pour doter la ville d’équipements structurants – piscines, salles de sport –, sera dans l’incapacité d’équilibrer son budget en 2025.

loi, les communes qui se regroupent au sein d’un établissement public de coopération communale peuvent gérer en commun des équipements ou des services publics et élaborer des projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la commune. Pour soutenir ce modèle, les EPCI à fiscalité propre disposent de la dynamique de fiscalité économique perçue sur le territoire de leurs communes membres. En contrepartie, ils reversent à leurs communes les attributions de compensation correspondant au montant des charges communales liées à l’exercice des compétences transférées à l’EPCI. Les attributions de compensation peuvent être révisées librement, à tout moment. publie un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice de ses compétences. Par ailleurs, la dotation de solidarité communautaire, qui est obligatoire pour les métropoles, a pour objet de réduire les disparités de ressources et de charges entre communes membres. Ce mécanisme de péréquation tient compte de critères légaux obligatoires, comme le potentiel fiscal ou financier, et de critères complémentaires au choix de l’EPCI, cette dotation pouvant être révisée à tout moment selon les besoins de l’intercommunalité. les communes contribuant particulièrement à l’attractivité économique et au développement de leur métropole bénéficient en retour, comme toutes les communes membres, des infrastructures et projets conduits à l’échelon communautaire. Le Gouvernement estime que les dispositifs actuels – attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire – offrent une large latitude aux collectivités membres d’une intercommunalité pour s’entendre sur le partage des recettes de fiscalité économique et pour développer en commun les services publics de proximité répondant aux besoins de leur

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit, dans son article 7 pour le volet fiscal et dans son article 36 pour le volet budgétaire, de réformer le financement du compte d’affectation spéciale

ainsi que l’enfouissement de ces derniers à des fins de résilience. En la matière, il nous faut envisager que l’exceptionnel dure. Or la réforme prévue dans ce projet de loi de finances remplace la contribution versée par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité par une fraction de l’accise sur l’électricité. Les syndicats d’électricité soulignent que cette réforme reposerait sur un tarif uniforme dans le pays, au détriment de la solidarité territoriale et de la nécessaire péréquation entre territoires urbains et ruraux. d’accise serait de plus décorrélée des besoins d’investissement constatés sur le terrain. Nous devons enfin craindre, à terme, la fin de ce compte spécial et la dilution des crédits liés à des missions de service public dans le budget de l’État.

ministre délégué. Monsieur le sénateur Roux, vous l’avez dit, le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, le Facé, est un outil indispensable pour soutenir les investissements dans les réseaux électriques des territoires ruraux, au bénéfice des collectivités et des populations. Il constitue un levier déterminant en faveur de l’égalité des territoires. Le Facé est nécessaire à l’action des collectivités qui concourent à la résilience des réseaux de distribution, au maintien de la qualité de la distribution et à la dynamique en faveur de la transition énergétique. Désormais, l’électrification de nouveaux usages et le raccordement de nouvelles productions d’énergie renouvelable solliciteront davantage les réseaux électriques et nécessiteront leur renforcement.

au sous programme d’investissement faisant l’objet d’une répartition départementale, a dû être reventilée en 2024 afin d’accompagner les dégâts causés par les tempêtes Ciarán et Domingos.

Nos priorités ne sont pas celles d’une moitié de la France contre l’autre moitié, mais celles de tous les Français. » Tous les Français ? Permettez moi d’en douter, monsieur le ministre. Comme Comme toujours, les outre mer sont les enfants oubliés de la République. Nos priorités sont vaguement écoutées à l’occasion de visites ministérielles éclair dans nos territoires. Elles sont entendues seulement quand le peuple, comme actuellement en Martinique, descend dans la rue pour manifester son mécontentement. Les Ultramarins, disait Aimé Césaire, sont des citoyens « entièrement à Que dire de mes compatriotes des zones enclavées de Guyane qui, chaque jour, constatent avec amertume que la République ne pense jamais à eux ? Une commune guyanaise sur trois n’est pas reliée au littoral par la route, monsieur le ministre. Près de 60 000 habitants ne peuvent compter que sur la pirogue pour se rendre dans une grande ville lorsque les avions sont cloués au sol. Ces déplacements sont pourtant obligatoires pour se soigner, pour suivre une formation ou tout simplement pour des raisons économiques. En 500 ans de présence en Guyane, la République n’a construit que

plus de 1 milliard d’euros pour une route de douze kilomètres à La Réunion ? Que doivent penser mes compatriotes quand l’État refuse d’augmenter sa participation à la continuité territoriale interne aérienne afin de permettre aux Guyanais de circuler

ministre délégué. Madame la sénatrice Phinera Horth, vous appelez l’attention du Gouvernement sur la situation des transports en Guyane, et plus largement dans l’ensemble des territoires ultramarins. Ces territoires sont au cœur de la politique conduite par le Gouvernement. raison pour laquelle le Premier ministre a souhaité que le ministre chargé des outre mer, François Noël Buffet, lui soit directement rattaché afin de coordonner au mieux l’action de tous les services de l’État en faveur de nos concitoyens ultramarins.

Le contrat de convergence et de transformation 2024 2027 prévoit la mobilisation par l’État de 171 millions d’euros de crédits, sur un total de 175,6 millions d’euros. cadre, quelque 152,4 millions d’euros seront consacrés à l’entretien et à la modernisation du réseau routier, dont plus de 100 millions d’euros financés exclusivement par l’État pour poursuivre l’aménagement de la route nationale 1. Le détail de ces opérations et de leur financement est en cours de discussion sous l’égide du préfet avec l’ensemble des élus locaux et des services mobilisés. La parole

comme l’une des plus accidentogènes de France. Les accidents souvent mortels étant de plus en plus nombreux, nous avons plaidé en 2017 pour une véritable accélération du chantier qui permettra la mise à deux fois deux voies des tronçons nord et sud de cette route en Saône et Loire. Grâce à la mobilisation de tous les élus locaux et avec le soutien de mes collègues parlementaires, en particulier

portant leur contribution totale à 126 millions d’euros pour une route nationale, dont je rappelle qu’elle relève de la compétence de l’État, monsieur le ministre. En 2021, un dépassement d’enveloppe dû à la révision des prix des matériaux et à des aléas a été révélé. Un nouvel effort de 12 millions d’euros a été consenti par le département et la région afin que les délais de travaux de la deuxième tranche soient tenus et que l’aménagement de cette infrastructure ne prenne pas de retard. Or nous apprenons que l’État, maître d’ouvrage de l’opération, envisage un échelonnement de la fin de cette deuxième tranche sur quatre ans, des travaux estimée au mieux en 2029, au lieu de 2025. Si cette information se confirmait, elle serait tout à fait choquante et inacceptable. Dans ce dossier, l’État doit être au rendez vous

des six sections aménagées seront terminées dans les mois à venir. Les deux dernières sections seront engagées en 2026 pour la section comprise entre La Fourche et le col des Vaux et achevées la même année pour la section Clermain Sainte Cécile.

Je vous remercie

ces 15 millions d’euros représentaient seulement 0,75 % du budget global du projet et avaient pour objectif de couvrir 7,5 kilomètres du tracé, sur un total de 32

Aucune réponse n’a été apportée à cette sollicitation. Pis, en juillet 2022, une réunion avec le préfet de région portant sur les mesures de protection acoustique a été annulée à la dernière minute sans aucune explication ; elle n’a jamais été reprogrammée. Quel mépris à l’égard des élus, des riverains et de l’association de défense qui les représente

ministre délégué. Madame la sénatrice Margaté, le Gouvernement soutient fortement la réalisation du CDG Express, qui est un projet indispensable pour améliorer la liaison entre le centre de Paris et son principal aéroport, Paris Charles de Gaulle.

des contraintes techniques, juridiques et financières applicables au projet. En ce qui concerne la tarification, il convient de rappeler que le projet CDG Express est financé sans subvention publique, dans le cadre d’un montage spécifique reposant notamment sur une concession de l’État dont les ressources proviennent d’une taxe appliquée sur les passagers aériens et d’une partie du produit des ventes des billets par l’exploitation du service ferroviaire, avec un tarif fixé spécifiquement pour la liaison. Je rappelle que cette ligne, dont les

Ces travaux coûteux, longs et nuisibles d’un point de vue environnemental sont prévus pour durer au moins neuf ans. Ils devraient émettre 30 000 tonnes de CO2, pour un coût de 1 milliard d’euros. Au delà de ces éléments connus depuis le démarrage du projet, l’inutilité publique de ces aménagements est désormais établie par le graphique de circulation S4 produit en 2023 par SNCF Réseau. Celui ci démontre la capacité des deux voies existantes à absorber tout le trafic prévu par le dossier de l’enquête publique préalable à la mise en service des lignes à grande vitesse (LGV), Bordeaux Toulouse et Bordeaux Dax, d’une part, et du RER métropolitain, d’autre part. Ce dossier prévoit jusqu’à huit trains par heure, alors que le graphique indique une capacité de dix trains sur les deux voies actuelles, et partant, une réserve de capacité de 25 %.

Enfin, j’insiste sur les conséquences, pour les riverains, des nuisances sonores liées à ces aménagements, en particulier à Bègles, où un ouvrage de type saut de mouton est prévu sans dispositif de protection phonique associé.

vous évoquez notamment le saut de mouton situé à Bègles. Une étude conduite par SNCF Réseau démontre que les niveaux de bruit réglementaires sont respectés sans protection acoustique. Pour autant, SNCF Réseau a pris en compte les remarques soulevées lors de l’enquête publique et réalisera les aménagements nécessaires à une diminution du bruit en construisant une corniche d’un mètre de haut.

Les récentes projections de circulation ferroviaire, en particulier liées au service express régional métropolitain (Serm) girondin, confirment la nécessité d’un tel projet. Aujourd’hui, quinze trains circulent dans les deux sens durant les deux heures de pointe du matin

Revitalisation fusionne les précédents zonages de soutien aux territoires ruraux, à savoir les zones de revitalisation rurale, les bassins d’emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural.

qui a été couronnée de succès : Gabriel Attal, alors Premier ministre, a ainsi annoncé le 4 juin 2024 que « ces 2 200 communes continueront […] à bénéficier des exonérations fiscales et sociales dont elles bénéficient actuellement. Cela vaut pour les commerces déjà en place comme pour les commerces qui s’installeront à l’avenir », ajoutant

répond à un objectif de simplification et d’efficacité des dispositifs de soutien aux territoires ruraux. Près de 17 700 communes ont intégré le nouveau zonage FRR. Attentif à l’attachement des populations et des élus des territoires concernés aux politiques de soutien, le Gouvernement a annoncé le 4 juin dernier que les quelque 2 200 communes situées en ZRR,

Conformément à cette décision, et afin de garantir son applicabilité, le Gouvernement propose, à l’article 27 du projet de loi de finances pour 2025, de faire bénéficier des effets du nouveau zonage FRR les 2 168 communes anciennement situées en ZRR, mais n’ayant pas intégré les nouvelles zones au 1 juillet 2024.

Des mesures dérogatoires en matière de délibération des exonérations de fiscalité directe locale sont également prévues, afin de permettre, dès 2025, une application du dispositif FRR aux entreprises créées ou reprises dans ces communes à compter du 1 juillet 2024. À cet égard, les collectivités auront jusqu’au 28 février 2025 pour instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter des impositions établies au titre de 2025. Cette disposition, prévue

de l’amende SRU. Or de tels investissements permettent aux communes d’augmenter leur part de logements sociaux, notamment en cœur de ville, là où les bailleurs sociaux refusent souvent d’intervenir.

Ce mécanisme vise à encourager les communes déficitaires à soutenir les opérations concourant au développement de l’offre de logements sociaux, et donc au rattrapage de leur déficit. Néanmoins, ces dépenses ne peuvent être déduites lorsqu’elles sont directement supportées par la commune, qui reste propriétaire du bien.

Lors des discussions relatives à l’élaboration du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, les professionnels concernés avaient souhaité établir une définition commune. Selon les administrations centrales, la demande relative à cette mention relevait non du droit national,

Ces administrations vérifient que la demande remplit toutes les exigences de la réglementation européenne relatives aux volumes concernés et à l’importance économique de la mention.

de monter en puissance. Les collectivités territoriales comptent sur elle pour éviter les dépôts sauvages. Le but est également d’améliorer la circularité des produits, le réemploi des matériaux et le recyclage des déchets.

Enfin, comme le prévoit le cahier des charges de la filière, les éco organismes ont commencé à distribuer des primes pour les produits intégrant des matériaux issus de ressources renouvelables gérées durablement, dont le bois fait encore une fois partie. Ils ont été incités à amplifier ces primes

Si la Camargue est souvent connue pour ses emblématiques flamants roses, de nombreuses espèces végétales et animales risquent de disparaître, ainsi que des pans entiers de notre patrimoine historique et économique. Les activités humaines ancestrales comme l’élevage de taureaux et de chevaux, la production de sel, la riziculture et la viticulture, qui ont façonné cette région, se trouvent aujourd’hui en péril. Les marais salants au cœur de cet écosystème fragile risquent de s’assécher si rien n’est fait. Pourtant, des ouvrages de protection existent ; ils ne demandent qu’à être entretenus et renforcés pour préserver cette terre si précieuse. si précieuse. Pour les passionnés et défenseurs de cet environnement unique, il est impensable d’accepter qu’il soit l’objet d’une politique de repli et de renoncement face aux enjeux du changement climatique. La Camargue est le fruit de l’action humaine ; elle est vivante, riche, et doit absolument être protégée.

des activités économiques et culturelles qui y prospèrent depuis des générations ? La parole

en évaluant les biens concernés à court, à moyen et à long terme. Les aménagements historiques de la Camargue ont permis de fixer le trait de côte au XX siècle. Pourtant, seulement la moitié des enrochements ont démontré leur efficacité. vous avez évoqué le besoin d’une attention particulière à ceux ci, mais il faut rappeler que, dans certains cas, la réalisation d’ouvrages de protection a accentué latéralement le phénomène d’érosion côtière. La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte actuellement en cours de révision préconise l’abandon des logiques de lutte contre la mer, lutte contre la mer, au profit d’une gestion respectueuse de la biodiversité et des phénomènes hydrosédimentaires. En Camargue, le syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer élabore actuellement une stratégie interrégionale qui traitera des aléas d’érosion et de submersion. Un programme d’action sera ainsi décliné dans le prochain plan littoral. le prochain plan littoral. C’est dans ce cadre d’une stratégie locale de gestion intégrée de la bande côtière que doivent être étudiées les différentes options d’adaptation au changement climatique. Les collectivités territoriales sont d’ailleurs déjà prêtes à faire évoluer leur politique d’aménagement, comme au Grau du Roi.

outre, le parc naturel régional de Camargue et l’État ont lancé une démarche participative pour élaborer une feuille de route avec l’objectif de faire face aux défis liés au sel et au changement climatique.

en l’occurrence de la région Île de France, soit seule comptable de l’artificialisation qui en résulte. De même, une communauté de communes accueillant un parc d’activités dont le rayonnement dépassera ses propres frontières, au bénéfice de toutes les

pour satisfaire leurs propres besoins de développement. La législation et la réglementation doivent donc tenir compte de ces artificialisations externes, au risque de laisser se créer de forts déséquilibres régionaux et de voir les territoires les plus dynamiques atteindre leurs objectifs de lutte

communales et intercommunales les zones artificialisées dans l’intérêt de plusieurs collectivités et de les imputer sur des enveloppes régionales, voire nationales.

et à quelques unes issues de l’inventaire du réseau partenarial des données sur les zones humides est tout à fait insuffisant, si ce n’est dangereux. Le système Ramsar fonctionne justement, car il a été imaginé indépendamment de toute mesure extérieure. Pourquoi chercher à abîmer cet outil, dont l’efficacité n’est plus à prouver en refusant un zonage étendu des BCAE 2 ? Il est urgent d’agir en faveur de ces zones, mais aussi de faciliter le dialogue entre l’administration et les particuliers. À partir du moment où les zones Ramsar seront liées dans l’esprit de tous, et notamment des agriculteurs concernés, aux BCAE 2, ces dernières y perdront énormément en termes d’image. Le choix qui a été fait d’une définition minimale du zonage des BCAE 2 n’est donc pas responsable en matière environnementale. Il ne répond pas non plus aux attentes de la profession agricole Madame la ministre, alors Monsieur le sénateur Michaël Weber, la France métropolitaine et les territoires vulnérables accueillent 30 % des espèces rares ou menacées, soit la totalité des amphibiens, la moitié des oiseaux ou encore le tiers des espèces végétales remarquables.

concerne les conditions à respecter pour les agriculteurs travaillant sur les zones humides ou les tourbières, la programmation 2023 2027 de la politique agricole commune impose, au 1 janvier 2025, la mise en place d’un zonage spécifique.

effectives et des tourbières. La BCAE 2 interdira les nouveaux remblais et réseaux de drainage pour préserver les sols existants, mais elle permettra également le maintien en l’état des réseaux de drainage.

très attaché au maintien des services publics de proximité dans nos territoires. Je tiens à vous rassurer : ce gouvernement ne souhaite en aucun cas réduire les services publics de proximité.

au titre de la loi n° 2022 229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis. Cette loi prévoit légitimement la réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. application de cette loi, les harkis ou les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et leurs familles ayant séjourné dans une ou plusieurs structures d’accueil entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, peuvent constituer un dossier auprès de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) pour obtenir une indemnité. Selon Selon le gouvernement de l’époque, plus de 50 000 personnes devaient ainsi pouvoir bénéficier de cette indemnisation. De nombreux harkis ont manifesté leur volonté de débuter ce processus de réparation : selon le bilan

elles ont été traitées et 16 000 ont reçu une réponse favorable, pour une indemnisation moyenne de 8 093 euros par dossier.

La séance est suspendue.

Merci